concernant l'attribution de la carte du combattant aux militaires présents sur le territoire algérien au-delà du 2 juillet 1962 soit enfin mise en oeuvre. Voilà enfin réparée la principale injustice qui altérait notre politique de reconnaissance envers nos anciens combattants s'agit, avec la revalorisation de l'allocation de reconnaissance en faveur des harkis, de l'un des rares motifs de satisfaction que nous réserve le projet de budget pour 2019. Rare, mais précieux, si bien que, malgré de nombreux points plus inquiétants, la commission des finances vous proposera néanmoins d'adopter les crédits de cette mission. Parmi nos inquiétudes figure la répétition de certains constats relatifs à la Journée défense et citoyenneté,

se tient toujours trop loin de ce que devrait être la vocation d'une journée consacrée à la défense de notre pays. Il faut espérer que le futur service national universel, le SNU, ne répétera pas les mêmes erreurs et qu'à cette occasion les difficultés rencontrées par une fraction importante de la jeunesse pourront être mieux prises en compte par les services de l'État. Le centenaire de la Grande Guerre s'achève. Malgré quelques couacs, je salue une commémoration qui a su être digne et participative dans beaucoup de

flamme, coeur et passion nos actions de mémoire, même les plus modestes. Les crédits consacrés à la reconnaissance de la Nation connaissent une baisse considérable.

plafonnement à 0,7 % de la revalorisation du point de pension militaire d'invalidité et, avec lui, de toutes les allocations qui en dépendent. La retraite du combattant ne bénéficie d'aucune amélioration, alors que la mission dégage spontanément plus de 6 % d'économies. Nous le regrettons ! Madame la secrétaire d'État, vous avez annoncé la création d'une commission tripartite destinée à envisager les questions posées par la revalorisation des prestations la création d'une commission n'est pas toujours un bon signe, mais peut-être pourrez-vous indiquer au Sénat ce que seront son rôle et sa composition ? En toute hypothèse, un objectif de maintien de la valeur réelle des prestations s'impose, ce qui passera sans doute par un mécanisme alternatif au rapport constant. Les allocations de reconnaissance vont certes connaître un certain dynamisme avec l'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie- je l'ai évoqué Cette mesure devrait coûter près de 60 millions d'euros pour 50 000 bénéficiaires, dont 30 millions d'euros au titre des avantages fiscaux. Comme ces derniers ne sont pas identiques pour chaque bénéficiaire, il sera intéressant d'identifier la répartition des soutiens

Il en serait ainsi pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, les OPEX, décidée en 2015. La réduction des effectifs de l'ONAC-VG sera-t-elle compatible avec un traitement rapide des 50 000 demandes relatives à la présence prolongée en Algérie ?

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues, je suis chargée de vous présenter les principales observations de la commission des affaires sociales en remplacement de notre rapporteur pour avis Bruno Gilles, qui ne peut être présent ce matin. La baisse naturelle du nombre d'anciens combattants permet, comme chaque année, une économie substantielle sur les prestations de reconnaissance et de réparation. Cette marge de manoeuvre est en partie mobilisée pour des mesures qu'il convient de saluer. L'attribution de la carte du combattant aux soldats qui ont servi en Algérie entre 1962 et 1964 correspond à une demande ancienne et le Sénat avait adopté une proposition de loi en ce sens au printemps dernier. Je ne peux donc que m'en réjouir. De même, le plan en faveur des harkis est bienvenu. Ces mesures expliquent largement l'avis favorable donné par la commission des affaires sociales à l'adoption des crédits de la mission, Toutefois, le coût de ces mesures demeure largement inférieur aux économies permises par la démographie des anciens combattants. Une réflexion sur les autres demandes du monde combattant pourrait donc être menée ; la discussion des amendements permettra d'en évoquer quelques-unes. Je souhaiterais notamment que le Gouvernement puisse nous donner des précisions quant à la situation des anciens supplétifs de droit commun et pour lesquels un traitement individualisé a été annoncé.

Cela signifie-t-il, comme l'ont compris les associations, que ces personnes bénéficieront de l'allocation de reconnaissance ? Qu'en est-il des dossiers écartés ? Par ailleurs, je regrette la diminution des crédits dédiés à la politique de mémoire. Cette baisse est nettement plus forte que le simple effet de la fin des commémorations liées au centenaire de la Première Guerre mondiale. Selon mes calculs, confirmés par les services du ministère des armées, ce sont près de 2,8 millions d'euros d'économies qui seraient prévus. Cette baisse pourrait paraître négligeable au regard des crédits de la mission, mais elle pourrait remettre en question de nombreux projets éducatifs, alors que la transmission de la mémoire aux jeunes générations apparaît plus que jamais nécessaire. Enfin, le nouveau contrat d'objectifs et de moyens entre l'État et l'office national des anciens combattants et victimes de guerre n'a toujours pas été conclu, alors que le contrat actuel arrive à échéance. Il serait souhaitable que le Gouvernement nous donne des garanties quant aux moyens qui seront accordés à l'ONAC-VG pour continuer à mener à bien ses missions et quant au maintien de son réseau territorial. Je vous rappelle

nous sortons tout juste du cycle mémoriel de la Grande Guerre, qui nous a permis d'honorer la mémoire de toutes celles et de tous ceux, civils ou soldats, qui ont chèrement payé le prix de la liberté. Ces commémorations ont offert un temps de mémoire utile à la reconnaissance de la Nation, ainsi qu'à la transmission de valeurs aux jeunes générations à une époque où la cohésion sociale a besoin d'être renforcée. sens, la mission que nous examinons aujourd'hui, dont une partie des crédits a porté le cycle du centenaire, est fondamentale. Si nous refermons un grand volet de la politique mémorielle, comme en témoigne la baisse, logique, des crédits du programme 167, nous devons poursuivre le travail d'affermissement des liens entre la Nation et son armée, ce sur quoi nous aurons sans doute l'occasion de débattre dans la perspective du service national universel. En attendant, le budget total de la mission s'élève à 2,3 milliards d'euros, ce qui représente une baisse d'environ 160 millions par rapport à la dotation de 2018. Cette diminution s'explique essentiellement par la baisse démographique naturelle des différentes catégories de bénéficiaires des prestations relevant du programme de reconnaissance et de réparation. La mission permet donc de préserver intégralement les droits des anciens combattants, aux côtés de la dynamique des dépenses fiscales. En outre, le projet de loi de finances pour 2019 introduit, dans le prolongement des dispositions adoptées les années précédentes, deux nouvelles mesures, sur lesquelles je souhaiterais m'arrêter plus particulièrement. La première concerne l'extension du bénéfice de la carte du combattant aux militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1 juillet 1964.

qui rétablit l'égalité entre frères d'armes et que le Sénat a souvent portée. Madame la secrétaire d'État, vous avez été sensible à cette demande récurrente du monde combattant et je me réjouis de la voir enfin concrétisée. La seconde mesure sur laquelle je voudrais m'attarder concerne le renforcement de la politique de reconnaissance et de réparation envers les harkis, pour un montant d'environ 23 millions d'euros en 2019. Je souhaite saluer les dispositions nouvelles, émanant notamment du rapport du préfet Dominique Ceaux intitulé « Aux harkis, la patrie reconnaissante. Je pense bien sûr à la revalorisation de 400 euros de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère versées aux supplétifs, ainsi qu'à la mise en place d'un dispositif d'aide individualisé aux enfants de harkis les plus en difficulté. en difficulté. Afin de compléter cet objectif d'équité dans la reconnaissance et la réparation, le groupe du RDSE souhaiterait que le chantier de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires soit approfondi. Il serait notamment souhaitable d'élargir la liste des bénéficiaires du titre de reconnaissance de la Nation aux vétérans ayant participé aux programmes d'essais nucléaires français sur les sites du Sahara et de Polynésie française de 1960 à 1996. Enfin, je souhaiterais insister une nouvelle fois sur la responsabilité qui est la nôtre en matière de mémoire, celle de prévoir l'après-centenaire. C'est essentiel et des moyens devront être mobilisés Nous devons souligner la grande réussite des commémorations qui se sont déroulées entre 2014 et 2018, ce que j'ai personnellement constaté dans mon département, la Meuse. Nous devons poursuivre sur cet élan. À mon sens, l'inscription des sites mémoriels de la Grande Guerre au patrimoine de l'UNESCO, dont le dossier sera de nouveau soumis en 2021, serait un moyen

il y a quelques jours, beaucoup de nos compatriotes se sont déplacés sur des lieux de mémoire afin de rendre hommage à ceux qui ont payé un lourd tribut pour la patrie. Les visages des plus jeunes, comme des plus anciens, exprimaient leur fierté pour les poilus et les femmes qui les ont soutenus. Ensemble, ils ont fait de la France une nation libre et rayonnante.

À cette dernière question, je rappellerai simplement les mots de Chateaubriand : « Les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts ; les morts, au contraire, instruisent les vivants ». Voilà le défi qu'il nous appartient de relever pour la génération actuelle et celles ensuite. Les crédits alloués à cette mission diminuent une fois de plus : le budget pour 2019 s'élève ainsi, en crédits de paiement, à 2,3 milliards d'euros. Depuis 2012, les dépenses ont ainsi reculé de près de 900 millions ! Madame la secrétaire d'État, cette trajectoire de repli demeure regrettable. Si elle peut s'expliquer, naturellement, par la diminution du nombre de bénéficiaires, elle n'apporte pas suffisamment de réponses aux besoins de revalorisation significative du pouvoir d'achat. J'y reviendrai. Cette baisse se reflète dans le programme 167. Si les crédits ont été en augmentation l'année dernière en raison des besoins liés aux commémorations, une économie de 20 % est à noter pour 2019. Toutefois, j'ai conscience que l'effort ne doit pas reposer uniquement sur les deniers de l'État. Le devoir de commémoration est l'affaire de tous. Des initiatives locales méritent d'être développées. Je pense notamment au département de l'Essonne, un drapeau à chaque commune pour que les enfants puissent le porter lors des cérémonies. Mais revenons au sujet principal ! Une exception demeure pour le financement de l'action Liens armée-jeunesse, qui connaît une progression de plus de 3 millions d'euros. voit en effet son périmètre élargi et prend désormais en charge une partie des financements du service militaire volontaire. C'est là un dispositif dont je veux saluer les mérites. Quant à la Journée défense et citoyenneté, elle demeure insuffisante compte tenu des objectifs auxquels elle entend satisfaire. Il convient donc de la réformer en profondeur. À cet effet, le Président de la République s'est engagé à créer un service national universel. À ce stade, aucune mesure ne figure dans cette mission. Le lundi 19 novembre, le groupe de travail missionné sur ce sujet a remis son rapport. Nous nous interrogeons et nous souhaitons avoir des précisions sur ce point. En outre, le programme 169, qui représente près de 90 % de la mission, n'échappe pas à la règle. Ses crédits diminuent également, et ce, de façon la plus importante, comme nous l'observons depuis 2015. Cela s'explique par la baisse du nombre de bénéficiaires, en particulier de ceux ayant combattu durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi en Indochine et en Afrique du Nord. Il eût été préférable d'encourager une revalorisation significative de la pension militaire d'invalidité et de la retraite du combattant. L'intention du Gouvernement de réunir une commission tripartite pour envisager une revalorisation du point d'indice serait déjà un premier pas, qui s'inscrirait dans le bon sens.

Il serait souhaitable que les mesures de réinsertion, comme le bilan de compétences ou l'accès à des formations relatives aux nouveaux métiers de l'Internet ou aux emplois réservés, soient proposées de manière plus formelle et plus systématique à cette catégorie de personnel. Il serait intéressant que le Gouvernement se penche sur cette proposition. De manière plus générale, la situation des forces participant aux opérations de protection des Français contre les actions terroristes doit être mieux prise en compte, comme celle de nos militaires de la quatrième génération du feu engagés sur différents théâtres d'opérations extérieurs. À ce sujet, nous souhaiterions avoir des informations sur le projet de mémorial national à Paris. Par ailleurs, il serait souhaitable qu'une plaque commémorative soit également apposée sous l'Arc de Triomphe en hommage aux morts pour la France en opérations extérieures. En termes budgétaires, cela ne représenterait rien, mais le symbole serait très fort. Ensuite, il pourrait être envisagé d'étendre la médaille commémorative d'Indochine, en retenant le 1 octobre 1957 comme date officielle de la fin des hostilités.

Pour terminer sur ce programme, nous regrettons la baisse de la subvention accordée à l'ONAC-VG à hauteur de 400 000 euros. De plus, nous souhaitons que l'assise retenue soit départementale, et non régionale. Concernant le programme 158, il connaît une hausse de plus de 5,2 millions d'euros. Cette augmentation est expliquée par l'accroissement des indemnités prévues au titre des spoliations antisémites. Par le biais de cette participation financière, la France s'honore. Mes chers collègues, encore aujourd'hui, nous devons rester vigilants. Comme toutes les formes de haine, l'antisémitisme doit être combattu sans relâche et avec la plus grande fermeté. Très Enfin, je terminerai par l'article 73, rattaché à la mission. Nous saluons la revalorisation de 400 euros de l'allocation de reconnaissance pour les harkis et de l'allocation viagère des conjoints survivants. Il s'agit d'un épisode de leur vie qui a été particulièrement douloureux. Ils ont combattu pour notre drapeau, pour la France. En conclusion, des avancées figurent dans ce projet de loi de finances. D'autres demandes sont à prendre en compte. Je sais pouvoir compter, madame la secrétaire d'État, sur votre sens de l'écoute-il est d'ailleurs très agréable de travailler avec vous.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les crédits consacrés aux anciens combattants. Alors que se terminent les célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale, la dette que la Nation entretient à l'égard de ceux qui ont versé leur sang hier et aujourd'hui apparaît plus vivace que jamais. Je veux rendre hommage à nos vétérans et à leurs familles de métropole et d'outre-mer pour les sacrifices consentis à la défense de la France. La patrie leur en est reconnaissante. Les Français n'oublient pas ce qu'ils leur doivent. Il nous semble néanmoins que la reconnaissance de la Nation ne doit pas seulement être un voeu pieux ou une incantation. Elle doit être une action concrète au service de nos soldats, une contribution collective à leur bien-être et à celui de leur famille. Si la diminution des crédits pour 2019 s'explique en partie par la baisse naturelle du nombre de bénéficiaires des différents dispositifs, nous serons vigilants à ce que cette baisse tendancielle ne représente pas un déclin des conditions de reconnaissance de la Nation. Vous nous rassurez sur plusieurs points, madame la secrétaire d'État. Vous avez pris des mesures fortes pour corriger des inégalités connues de longue date. Il s'agit, par exemple, de la revalorisation substantielle- 400 euros -de l'allocation de reconnaissance versée aux supplétifs de l'armée française en Algérie. Il s'agit également des mesures en faveur des enfants de harkis. Il s'agit enfin d'une mesure que nous avons longtemps attendue : l'octroi de la carte du combattant aux soldats présents sur le territoire algérien entre le 2 juillet 1962 et le 1 juillet 1964. Ces mesures sont autant de promesses tenues que nous saluons, comme nous saluons, madame la secrétaire d'État, votre volonté de passer en revue l'ensemble des questions en suspens avec le monde des anciens combattants. Nous espérons que la concertation annoncée portera davantage de fruits à l'avenir. Toutefois, malgré ces avancées, des injustices persistent et on peut noter la relative timidité de ce projet de budget, notamment la très faible revalorisation des pensions militaires d'invalidité.

trop peu connu en métropole, mais qui fait des merveilles pour l'emploi des jeunes en outre-mer. Je pense également à l'érection du monument pour les opérations extérieures, qui permettra aux citoyens de rendre hommage aux soldats tombés pour leur défense. Toutes ces initiatives sont bienvenues. Néanmoins, il ne doit pas être uniquement question de moyens budgétaires ou humains, car il s'agit au fond de réfléchir à ce qui fait de nous une nation, les valeurs justifient le combat, les blessures et le sacrifice ultime de nos soldats. Il s'agit, enfin, de mettre nos politiques de mémoire au service de l'avenir et d'un véritable projet de société par la transmission et le partage. Nous attendons donc avec impatience que se précise l'architecture du futur service national universel et, surtout, que soient enfin définies les modalités de son financement. Dans cette attente, le groupe Les Indépendants votera, en signe d'encouragement,

Cette paix, c'est l'héritage qu'ils nous offrent et c'est celui que nous devons laisser aux citoyens de demain, alors que l'extrême droite- le fascisme parfois -se réinstalle tout doucement dans le monde, en Europe en particulier. C'est là que réside le devoir de notre pays, le devoir de mémoire, que nous devons mener avec des moyens considérables, car si Alfred de Musset ne badinait pas avec l'amour, nous, parlementaires, ministres, élus locaux ou nationaux, ne badinons pas avec la haine. Soyons intransigeants face au racisme et au rejet de l'autre ! Je crois que les nombreuses commémorations du centenaire qui viennent de s'achever

visant à attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les accords d'Évian, du 2 juillet 1962 jusqu'au 1 juillet 1964.

Si nous pouvons nous féliciter des deux avancées majeures que je viens de citer, j'estime, en tant que femme, que nous devons également réparer une inégalité qui perdure depuis des années : je veux parler de la demi-part fiscale des veuves des anciens combattants.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je souhaite aujourd'hui porter la voix des associations représentatives du monde combattant, qui ont toute ma considération et dont j'ai plaisir à rencontrer les représentants locaux, tout au long de l'année, dans mon département, le Calvados. Ces associations ne se contentent pas d'agir pour le droit à réparation et le devoir de mémoire, elles participent aussi et surtout activement à la vie de la cité, sous des formes diverses. Gardiennes des valeurs qui fondent notre République, elles contribuent à réunir des personnes de toutes conditions autour d'actions caritatives, d'événements patriotiques ou concourant aux bonnes relations internationales. En cela, elles constituent assurément de merveilleux outils d'intégration et de cohésion sociale. Le budget pour 2019 de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » s'établit à 2,3 milliards d'euros. Ses crédits connaissent une forte diminution, de près de 160 millions d'euros, principalement liée, il est vrai, à la baisse du nombre des bénéficiaires des dispositifs de reconnaissance et de réparation. Il est néanmoins regrettable que le Gouvernement n'ait pas fait le choix, en dehors de certaines mesures, de redéployer les économies réalisées pour améliorer, à budget constant, les dispositifs existants. Cette mission regroupe trois programmes de poids financier très inégal. Le programme 167, qui représente 5 % des crédits de la mission, finance la Journée défense et citoyenneté, ainsi que les actions éducatives et mémorielles. Mon groupe est particulièrement attaché à tout ce qui peut concourir à l'exercice du devoir

pour assurer leur droit à vivre libres, égaux et dans la fraternité. De ce point de vue, il est particulièrement positif que le monument à la mémoire des soldats tombés en opérations extérieures puisse enfin voir le jour. Je sais qu'il est très attendu par nos jeunes anciens combattants et nos militaires actuellement engagés dans les conflits. les conflits. Je note aussi avec satisfaction que les commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale se sont bien déroulées. Les manifestations étaient particulièrement dignes, émouvantes et participatives : une réussite permise, comme toujours, grâce au dévouement de nombreux bénévoles.

près de 2,8 millions d'euros d'économies sont prévus, soit 20 % des crédits votés pour 2018. Là aussi, c'est regrettable, à une époque où la transmission de la mémoire, l'affirmation des liens entre la Nation et son armée sont véritablement nécessaires. Ce sont nos associations représentatives du monde combattant, sur le terrain, qui pourraient directement en pâtir, ainsi que nos jeunes, avec la remise en cause de certaines actions éducatives.

De nombreux événements, dont la cérémonie commémorative internationale en présence de chefs d'État, seront organisés, dans le Calvados notamment. Les coupes dans les lignes budgétaires dédiées à la mémoire ou à la nécessaire rénovation des sépultures apparaissent donc clairement excessives. Pour en terminer avec ce programme, j'indique que la commission des affaires sociales a été alertée sur le fait qu'aucun crédit n'était prévu pour le financement du service national universel, appelé à remplacer la Journée défense et citoyenneté. Il ne faudrait pas que les crédits de la mission soient ponctionnés en cours d'exercice pour financer ce nouveau dispositif.

le Gouvernement ait confirmé l'attribution de la carte du combattant aux soldats ayant servi en Algérie entre juillet 1962 et juillet 1964. Il s'agit d'une revendication ancienne du monde combattant, plusieurs fois relayée au Sénat, par moi-même comme par mes collègues, notamment en juin dernier au travers de l'adoption d'une proposition de loi visant à la satisfaire. À terme, cette mesure pourrait profiter à près de 50 000 personnes. Dès cette année, l'inscription budgétaire s'élèvera à 6,6 millions d'euros. Autre mesure annoncée, la revalorisation des expertises médicales nécessaires en vue de l'attribution de pensions militaires d'invalidité : j'espère que cela permettra de réduire les délais actuels, très difficilement supportables pour nos anciens. J'en viens à l'article 73 et aux conclusions du groupe de travail sur la situation des harkis, qui ont conduit à la prise de mesures nouvelles allant dans le bon sens : la revalorisation de 400 euros de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère et l'institution d'un dispositif de solidarité au profit des descendants des harkis. de 2019, 10 millions d'euros sont inscrits pour compléter les mesures en faveur des harkis et de leurs enfants. Si ces différentes mesures sont à souligner et à saluer, leur financement ne représente qu'une fraction réduite des économies permises par la baisse du nombre d'anciens combattants et, dans les faits, plusieurs demandes des associations représentatives du monde combattant sont toujours insatisfaites. Je citerai notamment le droit à l'indemnisation pour les pupilles de la Nation dont les parents ont été reconnus « morts pour la France » entre 1939 et 1945. Je fais ainsi le lien avec le programme 158, qui permettra, l'an prochain, de financer à hauteur de 106 millions d'euros différentes indemnités accordées aux victimes d'actes de barbarie et de persécutions commis pendant l'Occupation.

J'ai été particulièrement alertée sur la situation financière de nombreuses femmes, qui subissent une chute de revenus énorme après le décès de leur mari, au point de se retrouver dans un extrême dénuement. Ce n'est pas acceptable

en OPEX. L'ONAC-VG poursuit sa modernisation, mais celle-ci doit se faire en préservant les indispensables liens de proximité tissés avec les bénéficiaires et associations locales représentatives du monde combattant. Il faut conserver le maillage départemental de l'ONAC-VG et peut-être mieux harmoniser les pratiques entre territoires.

En cette année du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, je ne saurais conclure sans avoir une pensée pour tous ceux qui ont combattu pour défendre notre patrie. Que leur souvenir guide nos actions ! Très bien

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la mission interministérielle « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » constitue un trait d'union entre la société civile et le monde combattant, ainsi qu'entre les générations. En ma qualité de vice-présidente du groupe d'étude des sénateurs anciens combattants et de la mémoire combattante, je voudrais souligner tout son intérêt. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui se sont mobilisés autour des commémorations de la Grande Guerre et saluer les nombreuses initiatives prises à travers toute la France. Au nom du groupe Les Républicains, je souhaite en cet instant témoigner notre reconnaissance à l'ensemble du monde combattant, aux associations et à leurs bénévoles : nous savons combien leur travail est inestimable. veux également rendre un hommage solennel aux soldats français, qu'ils se trouvent sur le sol national, en OPEX ou en mer : ils sont les anciens combattants de demain. Depuis cet hémicycle, nous les assurons de notre soutien indéfectible. Nous pensons également à leurs familles, qui payent quotidiennement un lourd tribut à la défense nationale. Depuis 2007, 154 soldats sont morts en OPEX. Si l'on peut se réjouir de la mise en place de la Direction du service national et de la jeunesse, qui est chargée de la coordination de l'ensemble des initiatives ministérielles en matière de jeunesse, je voudrais appeler l'attention sur les classes « option défense et sécurité globales mises en place dans les territoires en partenariat avec les acteurs locaux. Cet enseignement suscite un réel engouement parmi les élèves, comme en témoigne le succès rencontré par l'expérience menée, dans mon département des Hautes-Alpes, à la cité mixte d'Embrun. C'est pourquoi je souhaiterais que les missions de la DSNJ soient élargies afin que cet enseignement facultatif soit mieux accompagné et, surtout, mieux valorisé. égard aux menaces qui pèsent sur notre pays, il est essentiel de promouvoir l'esprit de défense et de cohésion nationale. Madame la secrétaire d'État, pays rassemblé rime avec mémoire apaisée

à revoir les dossiers des anciens supplétifs, encore et toujours bloqués du fait des différentes jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation. Il est temps de clore ce chapitre avec la dignité qui s'impose. Tel est le sens de l'un de nos amendements. Depuis quelques années maintenant, l'Institution nationale des invalides, l'INI, connaît une modernisation. Pour les élus du groupe Les Républicains, cette institution est la maison des invalides de guerre. Elle doit le rester, et même devenir plus attractive plus qu'un symbole pour les soldats, c'est un lieu de mémoire vivante autant qu'un lieu d'hommage, témoignant du sacrifice physique et mental consenti par les soldats français pour leur pays. Depuis 2007, 620 soldats ont été blessés en OPEX. Enfin, madame la secrétaire d'État, je souhaite attirer votre attention sur un sujet important, celui des conséquences du désengagement de l'État de la Française des jeux. La loterie nationale a été créée en 1933 afin de financer les besoins des « gueules cassées

Pour conclure, nous comprenons que les crédits connaissent une baisse, pour des raisons inhérentes à la logique démographique. Néanmoins, nous voulons solennellement dire ici que cela ne pourra pas toujours justifier la poursuite d'une tendance baissière,

Monsieur le président, madame le secrétaire d'État, chers collègues, mes parents étaient instituteurs dans un petit village du Pas-de-Calais, sur ces collines de l'Artois où les batailles meurtrières de la Première Guerre mondiale ont couvert de cimetières toutes les terres environnantes. Enfant, j'ai assisté à toutes les commémorations patriotiques qui avaient lieu dans la cour de l'école, où nous habitions. Ces souvenirs sont ceux d'un enfant qui a trouvé son ancrage dans les valeurs républicaines au contact des anciens qui se sont battus pour que nous puissions être libres. Aujourd'hui plus que jamais, je suis convaincue que la transmission aux nouvelles générations de l'histoire de notre pays est une vraie mission : mission d'hommage envers celles et ceux qui ont combattu au péril de leur vie ; mission d'évaluation des dangers, des alliances, des pressions, des rancoeurs entre peuples, pour éviter que notre pays ne commette à nouveau les erreurs qui ont conduit à l'engrenage meurtrier.

et liens avec la Nation » du projet de loi de finances pour 2019 doit traduire en chiffres cette considération de la Nation. Des revendications portées de longue date par les anciens combattants et soutenues par le Sénat ont enfin été entendues par le Gouvernement.

L'an dernier encore, nous avions adopté un amendement au projet de loi de finances tendant à élargir les conditions d'attribution de la carte du combattant au bénéfice des membres des forces présentes en Algérie entre 1962 et 1964. Nous nous félicitons que le Gouvernement ait répondu favorablement à cette demande ancienne du Sénat. Je n'oublie pas non plus la revalorisation de 400 euros de l'allocation de reconnaissance en faveur des harkis, ainsi que la création d'un fonds pour les descendants de harkis en difficulté socioprofessionnelle. Cette reconnaissance me semble répondre à une injustice qui leur a été faite il y a maintenant bien longtemps. devoir de mémoire, 2018 a été une année historique de commémoration et de transmission. Si nous comprenons parfaitement que les crédits affectés l'année dernière à la célébration du centenaire

Nous avons un devoir de transmission à l'égard des jeunes. Connaître le passé est essentiel pour comprendre le présent. Pourtant, selon un sondage de CNN réalisé cette semaine en Europe, 24 % des jeunes Français de 18 à 34 ans ne savent pas ce qu'est l'Holocauste ! sur sept pays sondés, c'est en France que l'on ignore le plus ce que c'est : 8 % des Français déclarent même n'en avoir jamais entendu parler ... Incroyable ! Il y a en France une déperdition des connaissances historiques touchant à la question du génocide des juifs. À l'heure où l'antisémitisme progresse, où des circulent sur les réseaux sociaux et où de nombreux jeunes se radicalisent, je pense que le Gouvernement ne prend pas

En cela, la politique de mémoire est indispensable, madame le secrétaire d'État, et je regrette sincèrement cette baisse de crédits. Il faut resserrer le lien entre la patrie et notre jeune public.

Est-il bien approprié de faire de la prévention en matière de sécurité routière lors d'une journée destinée à sensibiliser nos jeunes aux enjeux de la défense ? Cette journée a perdu sa cohérence et on ne pourra pas faire l'économie

: La parole est à Mme Corinne Féret. Il s'agit, au travers de cet amendement, de financer une extension de l'indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. En 2000, le Gouvernement a reconnu le droit à indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et racistes pendant cette guerre. Dès la fin de 2001, le Gouvernement a été sollicité pour que d'autres orphelins de victimes de la barbarie nazie puissent bénéficier des mêmes indemnisations que les victimes de la Shoah.

il s'agit, au travers de cet amendement, de financer une extension du champ de l'indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Un consensus existe sur ce sujet au sein de la représentation nationale ; nous devons lui donner une

Dès la fin de 2001, le Gouvernement a été sollicité pour que d'autres orphelins de victimes de la barbarie nazie puissent bénéficier des mêmes indemnisations que les victimes de la Shoah.

Les victimes en question ont déjà pu bénéficier d'une certaine reconnaissance de la Nation. Par ailleurs, en l'état, il n'existe pas de base légale susceptible de fonder une indemnisation particulière, si bien que la portée de ces amendements est incertaine. Les coûts d'une telle indemnisation méritent d'être précisés ; on évoque parfois

les grands invalides de guerre, les conjoints survivants des morts au combat ou des grands invalides de guerre et les anciens combattants. La pension militaire d'invalidité indemnise le préjudice qui découle des blessures ou maladies ; la pension versée au conjoint survivant

Si, de cette manière, tous les préjudices des grands invalides de guerre ont été pris en compte et dignement réparés, il n'en a pas été de même pour les veuves de grands de grands invalides de guerre : le niveau de leurs pensions n'a pas évolué depuis 1928. Un véritable fossé s'est donc creusé entre le droit à réparation des grands invalides de guerre et celui de leurs conjoints survivants. Cette injustice s'est amplifiée au fil des ans. Les pouvoirs publics, récemment alertés par les associations, ont mis en place quelques dispositifs, mais les conditions requises sont toutefois si restrictives qu'à peine 10 % des veuves de grands invalides de guerre ont pu en bénéficier. Une grande partie des crédits votés n'ont donc pas été utilisés pour établir à un niveau décent le droit à réparation de nos veuves de guerre. Le présent amendement a pour objet de revaloriser la pension des conjoints survivants des grands invalides de guerre dont le niveau d'invalidité était supérieur à 100 % à la date du décès.

L. 111-2 du code du service national, « la Journée défense et citoyenneté a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre entre l'armée et la jeunesse ». L'article L. 114-2 du même code précise que la JDC est organisée pour tous les Français.

important. Le code du service national dispose que les Français établis hors de France doivent participer à la JDC, sous la responsabilité du chef de poste diplomatique et consulaire accrédité,

avez citée : on ne peut pas se soustraire à cette obligation législative. Pour tout vous dire, je suis particulièrement

II-3. Cet amendement, que je présente au nom de ma collègue Brigitte Micouleau, qui ne pouvait être présente ce matin, vise à corriger une discrimination persistante dans la reconnaissance par l'État des sacrifices consentis par les harkis. En effet, ceux-ci ne bénéficient pas du même traitement selon le statut juridique qui était le leur à l'époque Au côté de la très grande majorité des anciens supplétifs, qui relevaient du statut civil de droit local, des pieds noirs d'origine européenne, soumis au statut civil de droit commun, ont servi dans des formations supplétives comme des harkas, des sections administratives spécialisées ou des groupes mobiles de sécurité. Le bénéfice des mesures de réparation mises en place en faveur des anciens supplétifs, notamment l'allocation de reconnaissance, a toujours été réservé aux seuls harkis de statut civil de droit local. Toutefois, à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011, ce critère a été supprimé ; il n'a été rétabli que par la loi du 18 décembre 2013, dont la portée rétroactive a été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, le 16 février 2016. Dès lors, tous les anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui en ont fait la demande entre les mois de février 2011 et de décembre 2013 devraient mesures de réparation. Pourtant, l'administration a à l'époque « joué la montre » et refusé de répondre aux requêtes, afin de décourager tout recours contentieux. Ceux qui ont fait appel aux tribunaux ont depuis eu gain de cause. Il appartient maintenant d'agir au nom de celles et ceux qui n'ont pas pu le faire. Il s'agit d'une population âgée,

Cette mesure n'entraînera pas de dépense supplémentaire et est compensée par le déclin démographique du nombre de bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance, qui a diminué de 209 entre 2016 et 2017. Cet amendement vise donc, pour financer cette mesure, à procéder au

de loi de finances, notamment l'an dernier. À la suite de difficultés juridiques, certains anciens supplétifs de statut civil de droit commun se sont trouvés exclus du bénéfice de l'allocation de reconnaissance versée aux anciens supplétifs de statut civil de droit local.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le constat est partagé, je le crois, sur toutes les travées : depuis quelques années, le ministère de la justice n'a pas les moyens d'exercer convenablement ses missions. Les effets de l'augmentation de ses moyens intervenue ces dernières années tardent encore à se matérialiser. Dans les tribunaux ou les établissements pénitentiaires, les personnels expriment leurs difficultés à exercer leur métier, voire leur désarroi. En effet, la surpopulation carcérale ou des délais de jugement trop longs contribuent à décourager les agents, qui, parfois, ne trouvent plus de sens à leur action. C'est dans ce contexte de fortes attentes que s'inscrit ce projet de loi de finances : attentes en termes des moyens, mais aussi de fonctionnement même de la justice. À ce titre, le Gouvernement a présenté un projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, que le Sénat a largement amendé sur l'initiative de sa commission des lois. De véritables réformes sont en effet indispensables, car les moyens seuls ne suffiront pas au « redressement » de la justice, pour reprendre l'intitulé de la proposition de loi déposée par notre collègue Philippe Bas, président de la commission des lois. Madame la Madame la garde des sceaux, la commission des finances a émis un avis favorable sur l'adoption des crédits du ministère de la justice, considérant que l'augmentation de près de 4,5 % des crédits hors compte d'affectation spéciale « Pensions se justifie, s'agissant d'un ministère régalien que nous considérons comme prioritaire. Certains regrettent que la hausse des crédits ne soit pas plus importante. Je partage leur impatience, mais je pense que la proposition du Gouvernement est équilibrée. En effet, les hausses de crédits doivent être crédibles et il serait illusoire de penser pouvoir dépenser- judicieusement s'entend - beaucoup plus. En effet, une fois le budget voté, il faut l'exécuter, l'on se heurte alors à la réalité. Recruter et former du personnel, construire des établissements pénitentiaires, des juridictions, repenser des systèmes d'information : tout cela prend du temps et tous vos prédécesseurs, madame la garde des sceaux, en ont largement pris conscience. Lors de mes récents déplacements sur le terrain, j'ai eu l'impression que les choses commençaient, lentement, à s'améliorer, notamment dans les juridictions. Les vacances de postes semblent s'amenuiser, l'ouverture du nouveau palais de justice de Paris ou la réouverture prochaine de la prison de Paris-La Santé- sites que j'ai tous deux visités -sont des signes visibles que la situation commence à évoluer, même si le défi reste de taille. En ce qui concerne l'administration pénitentiaire, le projet de loi de finances prévoit une hausse de 95 millions d'euros des dépenses de personnel, afin notamment de créer de nouveaux postes de surveillant pénitentiaire pour combler les vacances. À cet égard, je souhaite vous poser quelques questions. Comment est-il envisagé de faire face à l'ouverture de nouveaux établissements pénitentiaires, conjuguée aux départs à la retraite et à des difficultés de recrutement de surveillants pénitentiaires ? pénitentiaires ? Pouvez-vous nous préciser les contours que devrait prendre la prime de fidélisation annoncée en janvier dernier à la suite du mouvement social de la fin de 2017 ? Combien d'agents seront concernés ? Quel en sera le coût ? Le programme de construction de nouvelles places de prison retenu par le Gouvernement est moins ambitieux que ce qu'avait initialement annoncé le candidat Emmanuel Macron. Il est pourtant urgent de garantir un encellulement individuel, mais aussi, tout simplement, de dignes conditions de détention, permettant aux surveillants d'accomplir convenablement leur travail. Le présent projet de loi de finances prévoit de consacrer près de 230 millions d'euros aux projets informatiques du ministère, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2018. Ces investissements sont le signe du rôle crucial que le numérique peut et doit jouer dans la modernisation de la justice. Il devra toutefois en résulter, à terme, des économies. La dématérialisation de la demande du bulletin n° 3 du casier judiciaire est une première étape, que je tiens à saluer, mais il faudra aller plus loin, en particulier en ce qui concerne les applications utilisées par le ministère lui-même, mais aussi avec ses partenaires, qu'il s'agisse des services de police ou de ceux Il conviendra de veiller à ce que la numérisation des procédures et des démarches demeure compatible avec un accès au droit sur l'ensemble du territoire, afin qu'à la fracture sociale et territoriale ne s'ajoute pas la fracture numérique. je tiens également à vous faire part d'une inquiétude concernant le dynamisme des frais de justice. Il est justifié que les magistrats souhaitent recourir à toutes les techniques modernes existantes en vue de la manifestation de la vérité et leurs décisions ne sauraient être contraintes par des questions de coûts. Si d'importants progrès ont déjà été réalisés pour rationaliser le circuit de la dépense, les charges à payer demeurent particulièrement élevées. Les crédits de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, augmentent, notamment afin de financer la création de cinq nouveaux centres éducatifs fermés.

Ainsi, elle est passée de 360 millions d'euros en 2015 à 507 millions d'euros en 2019, soit une augmentation de 41 %. L'aide juridictionnelle est financée en partie par des crédits budgétaires, en partie par des ressources fiscales affectées au Conseil national des barreaux. Dans ce contexte de croissance forte de l'aide juridictionnelle, une révision de ses modalités de financement paraît indispensable ; nous en reparlerons à l'occasion de l'examen des amendements.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, les crédits de la mission « Justice » progressent de 4,5 % en 2019, hors dépenses de pensions, pour atteindre un montant total de 7,29 milliards d'euros en crédits de paiement, identique à celui qui a été prévu par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de programmation 2018-2022

« Accès au droit et à la justice », « Conduite et pilotage de la politique de la justice » et « Conseil supérieur de la magistrature » augmentent quant à eux de 2,29 %, et leurs autorisations d'engagement de 2,94 %.

Le schéma de création d'emplois est plus ambitieux que l'année dernière, avec la création de 192 postes dans les juridictions judiciaires. Le nombre de postes vacants de magistrat a baissé de façon significative en 2018 : on ne compte plus que 252 vacances de postes de magistrat au 1 octobre 2018, contre 417 l'année précédente. Les crédits de paiement en matière d'investissement progressent de 8,5 % par rapport à 2018 et les autorisations d'engagement de 211 %, ce qui s'explique par le lancement d'un nouveau programme pluriannuel de rénovation et de construction dans l'immobilier judiciaire. Ce programme est très attendu, madame la garde des sceaux, étant donné le piètre état des locaux de trop nombreuses juridictions. En dernier les crédits en faveur de l'informatique et du numérique augmentent de 20 % entre 2018 et 2019. Ces mesures ne peuvent cependant pas occulter une situation qui demeure encore fragile dans les juridictions. Ainsi, les délais de traitement des affaires continuent de croître, tant en matière civile qu'en matière pénale. En matière civile, ils sont passés de 7,5 mois en 2007 à 11,8 mois en 2017 devant les tribunaux de grande instance, et de 12,7 mois à 14,7 mois devant les cours d'appel.

Les tribunaux de grande instance vont en outre devoir absorber, à compter du 1 janvier 2019, le contentieux social actuellement traité par les tribunaux des affaires sociales et les tribunaux du contentieux et de l'incapacité, suscite beaucoup d'interrogations parmi les personnels, madame la ministre. De même, les frais de justice demeurent une source d'inquiétude. Même s'ils font l'objet d'une meilleure budgétisation, leur augmentation est constante. Vous trouverez dans le rapport écrit quelques chiffres parlants, mes chers collègues. Pour terminer

Le Sénat a fait des propositions concrètes et utiles lors de l'examen du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Veuillez conclure. Il a notamment proposé le rétablissement d'une contribution à l'aide juridique en première instance et l'instauration de l'obligation de consultation préalable d'un avocat avant toute demande d'aide juridictionnelle. Le Gouvernement est resté sourd à ces propositions jusqu'à C'est pourtant un enjeu essentiel. Madame la garde des sceaux, que comptez-vous faire pour sauver un système qui est aujourd'hui à bout de souffle ? Au bénéfice de ces observations, et malgré ces fortes réserves, la commission des lois a donné un avis favorable à l'adoption des crédits des programmes de la mission « Justice » concernant la justice judiciaire et l'accès au droit. Monsieur le

mais cette hausse est insuffisante au regard des besoins de l'administration pénitentiaire et des enjeux du redressement de la justice. Pour l'administration pénitentiaire, 2018 a été une année de crise. Le début de l'année a été marqué par un important mouvement de contestation des surveillants pénitentiaires, qui sont aujourd'hui en nombre insuffisant pour faire face à la surpopulation carcérale. Ce mouvement a été suivi, au printemps, de la mobilisation des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui ne peuvent plus suivre correctement et efficacement les personnes condamnées en milieu ouvert. Au mois de juillet, une évasion spectaculaire, celle de Rédoine Faïd, a soulevé de nombreuses questions quant à la sécurité de nos établissements 2018 a été une année critique, de nouveaux records ayant été battus en matière de surpopulation carcérale : au 1octobre 2018, 70 714 personnes étaient détenues, soit 3,1 % de plus qu'un an auparavant. Actuellement, le taux d'occupation moyen de nos maisons d'arrêt est supérieur à 140 %. Imagine-t-on que des détenus puissent se réinsérer à leur sortie lorsqu'ils passent vingt heures par jour dans une cellule de 9 mètres carrés avec un ou plusieurs codétenus ?

à l'engagement présidentiel de construire 15 000 nouvelles places de prison sur le quinquennat. Le plan pénitentiaire que vous avez annoncé nous paraît insuffisant, voire trompeur à certains égards. Il est insuffisant, car il ne prévoit la livraison que de 7 000 places environ d'ici à 2022, dont un peu moins de 5 000 seulement concerneront les maisons d'arrêt et les centres pénitentiaires. Les 2 000 autres places sont destinées à des structures d'accompagnement vers la sortie, les SAS. Or, pour atteindre un taux d'encellulement individuel de 80 % en 2022, et au regard des trajectoires d'évolution de la population carcérale, il aurait fallu livrer au moins 9 500 nouvelles places de prison, en privilégiant les établissements pour peines. Lors de sa visite de la maison d'arrêt de Paris-La Santé, notre collègue Alain Marc a constaté avec effarement que toutes les cellules individuelles de 9 mètres carrés avaient d'ores et déjà été « doublées », des lits superposés ayant été installés afin de pouvoir y accueillir deux personnes dès la réouverture de l'établissement, au mois de janvier prochain.

avis. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, lors de sa réunion du 21 novembre dernier, la commission des lois a donné un avis favorable à l'adoption des crédits du programme « Protection judiciaire de la jeunesse » du projet de loi de finances pour 2019. La commission des lois a été sensible à l'effort consenti en faveur de la protection judiciaire de la jeunesse, dont les crédits augmentent de 2,8 %, pour atteindre 875 millions d'euros en 2019. Ces moyens supplémentaires permettront la création d'une cinquantaine de postes, principalement des emplois d'éducateur, mais aussi de psychologue et d'assistante sociale, et ils financeront des travaux de rénovation et d'entretien des locaux trop longtemps différés. Il faut aussi souligner l'effort consenti en faveur du secteur associatif habilité, dont les crédits vont être revalorisés afin de lui permettre de réaliser un plus grand nombre de mesures d'investigation. Une partie non négligeable des crédits supplémentaires alloués à la protection judiciaire de la jeunesse sera affectée à la construction de nouveaux centres éducatifs fermés, ou CEF. Le Gouvernement prévoit 1,8 million d'euros pour commencer les opérations nécessaires à l'ouverture de deux centres dans le secteur public et 2,3 millions d'euros pour faciliter le lancement de cinq CEF associatifs. Les auditions et les déplacements auxquels j'ai procédé n'ont pas levé toutes les interrogations concernant la construction de ces nouveaux CEF. J'ai entendu formuler de nombreuses questions concernant l'évaluation des besoins qui justifie l'ouverture de 240 places supplémentaires, alors que les cinquante-deux CEF aujourd'hui en activité sont loin d'être saturés. Les professionnels s'inquiètent de la concentration des moyens humains et financiers sur ce programme de construction. Je sais que vous êtes convaincue, madame la ministre, de la nécessité de préserver une palette diversifiée de modes de prise en charge, afin que les juges des enfants puissent trouver une solution adaptée à chaque jeune. Mais aurez-vous les moyens, dans les années qui viennent, de financer l'ouverture de vingt nouveaux CEF sans pénaliser les autres dispositifs de la protection judiciaire de la jeunesse ? Peut-être pourrez-vous nous préciser vos intentions dans la suite de ce débat. Pour conclure mon propos, j'évoquerai la réforme de l'ordonnance de 1945. La commission des lois y est favorable, cette ordonnance étant devenue peu lisible au fil de ses modifications successives et devant être adaptée à l'évolution de la délinquance juvénile. Cependant, nous ne pouvons que déplorer le choix du Gouvernement et de la majorité à l'Assemblée nationale de recourir à une ordonnance pour y procéder. Qui plus est, la demande d'habilitation a été introduite par voie d'amendement à l'Assemblée nationale lors de la discussion du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, que nous avons examiné en procédure accélérée au mois d'octobre. Je sais que vous prévoyez d'associer des parlementaires à l'élaboration de l'ordonnance, mais nous sommes nombreux à penser qu'une réforme d'un dispositif de cette importance mériterait un débat plus approfondi devant la représentation nationale. Mes chers collègues, je vous

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le budget de la mission « Justice » progresse de près de 4,5 %, pour atteindre 7,291 milliards d'euros en crédits de paiement. Même si le budget pour 2019 s'inscrit dans le mouvement de hausse quasiment continue des ressources votées, la trajectoire budgétaire retenue par le Gouvernement dans le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice-

est insuffisante pour assurer le redressement du service public de la justice par une action puissante et durable de rattrapage des retards accumulés dans le passé. Oui, cette progression de près de 4,5 % apparaît bien modeste au regard des efforts nécessaires au redressement de la justice, qui se trouve aujourd'hui dans une situation critique, en termes tant de délais que de moyens et Territoires l'avait déjà fait il y a un an à cette même tribune. Le rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, qui a été récemment publié, vient confirmer, hélas ! ce diagnostic

Je formulerai maintenant des observations spécifiques sur deux des trois programmes de la mission « Justice ». Concernant tout d'abord les crédits consacrés à la justice judiciaire et à l'accès au droit, si le projet de loi de finances pour 2019 comporte plusieurs mesures positives, celles-ci doivent toutefois être accueillies avec prudence et ne doivent pas occulter une situation qui demeure extrêmement dégradée dans les juridictions. Cette année encore, nous déplorons la pénurie chronique de magistrats et de fonctionnaires de greffe. Cette situation se traduit par un délai moyen de traitement des procédures en augmentation, toutes juridictions confondues. De même, le système de l'aide juridictionnelle est à bout de souffle. À cet égard, le Sénat avait proposé le rétablissement de la contribution pour l'aide juridique en première instance, modulable de 20 à 50 euros, et l'instauration de l'obligation de consultation préalable d'un avocat avant toute demande d'aide juridictionnelle. Concernant les crédits du programme « Administration pénitentiaire », je déplore l'hypocrisie de l'annonce du programme « 15 000 places », lequel repose essentiellement sur des constructions engagées par des gouvernements précédents. Ici, le constat est clair : le plan de construction de 15 000 places supplémentaires de prison d'ici à 2022 dont la mise en oeuvre figurait parmi les engagements de campagne du Président de la République a été abandonné. Les ambitions du Gouvernement ont été ramenées, pour l'essentiel, à la création de 2 130 places en structures d'accompagnement vers la sortie d'ici à 2022. Aucun chantier n'étant engagé à ce jour, tous les terrains n'ayant pas été identifiés, même cet objectif plus modeste risque fort de ne pas être atteint. Je souhaite également dénoncer l'insuffisance des crédits consacrés à la réinsertion, alors même que le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit de renforcer l'efficacité de l'exécution des peines.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, pour la deuxième année consécutive, vous nous présentez, madame la ministre, un budget pour la justice qui connaît une nouvelle progression de ses crédits. Après une hausse significative de 3,9 % en 2018, les crédits de la mission « Justice » augmentent à nouveau, de 4,5 %, soit 313 millions d'euros supplémentaires.

mais je tiens à souligner le volontarisme budgétaire du Gouvernement dans un contexte de redressement des finances publiques. Cela marque de façon évidente une volonté non feinte de placer la justice au rang des priorités gouvernementales. Cet effort financier notable vous permettra, madame la garde des sceaux, de mettre en oeuvre un engagement présidentiel important, inscrit dans le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice,

vous permettra de mener à bien les quatre chantiers prioritaires que vous vous êtes fixés : l'amélioration de la justice du quotidien ; le renforcement du sens et de l'efficacité des peines la diversification des modes de prise en charge des mineurs délinquants ; le renforcement de l'accès au droit et de l'aide aux victimes. Ces moyens permettront, entre autres choses, la mise en oeuvre du plan pénitentiaire que vous aviez présenté en septembre dernier et qui prévoit une évolution du parc pénitentiaire de notre pays, le renforcement de la sécurité des établissements pénitentiaires et la réinsertion des détenus.

Je profite d'ailleurs du temps qui m'est imparti pour attirer votre attention sur la situation des établissements pénitentiaires dans les outre-mer. En dépit d'améliorations récentes et en cours et de la création de nouvelles infrastructures, comme à Saint-Laurent-du-Maroni, l'état des prisons reste globalement déplorable dans ces territoires éloignés et présente des spécificités qui sont insuffisamment prises en compte, notamment s'agissant de la réinsertion des détenus. J'aurai l'occasion de revenir sur cette question lors de l'examen des crédits de la mission « Outre-mer », puisque j'ai souhaité en faire le fil directeur de mon avis. Madame

N'y a-t-il pas là une occasion de repenser l'organisation judiciaire au sein de ce département en difficulté et de le doter d'une cour d'appel de plein exercice ? Outre la reconnaissance supplémentaire de l'ancrage de Mayotte dans le droit commun des départements que cela induirait, il s'agit de permettre aux Mahorais d'accéder au service public de la justice comme tous les citoyens français.

À cet égard, l'importance des ressources dégagées en faveur du plan de transformation numérique- 97 millions d'euros et 80 emplois créés -mérite évidemment d'être soulignée. ce projet de budget de la justice pour 2019 est en adéquation avec les enjeux des réformes que vous souhaitez mener. Le groupe La République En Marche a déposé des amendements d'appel relatifs à l'aide juridictionnelle

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, un peu plus d'un mois après l'examen de la réforme de la justice, nous sommes aujourd'hui appelés à nous prononcer sur les crédits de la justice inscrits dans projet de loi de finances pour 2019. Sur les chiffres, je serai brève : la progression globale des crédits de 4,5 %, à 7,29 milliards d'euros, va à l'évidence dans le bon sens, bien qu'elle demeure insuffisante, eu égard au retard qu'a accumulé notre pays, pour assurer le redressement du service public de la justice. Les augmentations décidées année après année portent sur un budget historiquement si faible que le retard structurel n'est en effet jamais rattrapé, comme l'a d'ailleurs signalé la Commission européenne pour l'efficacité de la justice dans son rapport du 4 octobre 2018. Rappelons que la France dépense moins de 66 euros par an et par habitant

Or la philosophie de ce projet de budget nous inquiète au plus haut point : pour l'essentiel, les nouveaux crédits du programme « Protection judiciaire de la jeunesse » sont absorbés par la construction de vingt nouveaux centres éducatifs fermés, que le constat d'échec des cinquante-deux structures déjà existantes est établi, comme l'a récemment signifié une mission d'information sénatoriale sur la réinsertion des mineurs enfermés. Le caractère exceptionnel de l'enfermement des mineurs est pourtant déjà prévu par l'ordonnance la justice doit aller de pair avec l'éducation. L'enfermement devrait être relégué aux oubliettes de l'histoire. Nous connaissons déjà ses effets délétères sur les adultes, pourquoi persister à se fourvoyer en enfermant des mineurs ? ? Vous l'aurez compris, la progression des crédits de cette mission, qui fait de la Chancellerie un ministère prioritaire pour Bercy, ne saurait nous convaincre. Elle est trop faible pour permettre de rattraper le retard accumulé. Surtout, la ventilation des crédits augmentés est au service d'un projet de société et d'une vision de la justice

en raison de la surpopulation carcérale, les détenus souffrent d'une grande promiscuité, de conditions d'hygiène déplorables et de difficultés d'accès aux soins ainsi qu'au travail ou à la formation, ce qui exacerbe les violences, nuit à la réinsertion des personnes condamnées et explique, au moins en partie, le manque d'attractivité de la profession de surveillant pénitentiaire

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, depuis 2002, la mission « Justice » est devenue mission prioritaire du budget général de l'État. présent projet de loi de finances, un effort important, correspondant aux souhaits du Sénat, a été fait pour les crédits de la mission « Justice », à l'exception toutefois de ceux du programme « Administration pénitentiaire ». J'y reviendrai. La moyenne d'augmentation générale des autres programmes est satisfaisante. Seul le programme « Justice judiciaire » connaît une progression très inférieure. Du point de vue des financements accordés au fonctionnement des juridictions judiciaires, la France occupe en Europe un rang très médiocre la dépense par habitant s'élève à 65,90 euros par an, contre 122 euros en Allemagne, 119,20 euros aux Pays-Bas ou 75 euros en Italie. Notre rapporteur pour avis Yves Détraigne craint fort que, compte tenu de l'inflation, l'augmentation budgétaire de ce programme ne soit finalement que résiduelle Il recouvre pourtant l'ensemble des dépenses des juridictions judiciaires, le budget de l'École nationale des greffes- les greffiers sont les grands oubliés de la réforme -, la subvention versée à l'École nationale de la magistrature et le personnel affecté au sein du réseau judiciaire de proximité proximité est, elle aussi, passée en grande partie par pertes et profits. Certaines des juridictions transformées en chambres seront inévitablement fermées à l'avenir, madame la garde des sceaux, et ce sont encore les habitants des territoires ruraux qui en feront les frais. La question des moyens et de leur affectation est essentielle pour offrir à nos concitoyens une justice de qualité, une justice accessible offrant protection et garanties d'impartialité. Elle ne saurait en aucun cas trouver une solution dans de simples réorganisations, qui se révéleront à terme suppression de tribunaux d'instance, déjudiciarisation ou encore dématérialisation débridée des procédures. Comme les rapporteurs de la commission des lois, je constate que la trajectoire budgétaire retenue par le Gouvernement dans le projet de loi de programmation 2018-2022 est bien moins ambitieuse que celle proposée par le Sénat. Sera-t-elle suffisante pour redresser le service public de la justice ? Non, sauf à réduire drastiquement son rôle auprès des citoyens. Cela semble être le chemin pris

Je constate également que certaines ambitions du Gouvernement, reprenant les engagements de la campagne présidentielle, sont au mieux revues à la baisse, au pire abandonnées. Je veux bien sûr parler ici de notre politique pénitentiaire. Nous avons voté dès 2009 le principe de l'encellulement individuel. Près de dix ans plus tard, l'échec est patent. Les détenus sont parfois quatre par cellule, sans que l'administration ait même toujours la possibilité de les grouper par catégorie de faits commis. La douche des détenus entassés est loin d'être quotidienne, et je n'évoque pas les soins psychiatriques ... Inutile de souligner combien la réinsertion devient hasardeuse La situation des bâtiments est elle aussi profondément préoccupante. De nombreux établissements sont à la limite de l'insalubrité et leur sûreté n'est pas toujours garantie. Il avait été annoncé 15 000 places de prison supplémentaires en cinq ans ; le Gouvernement avance aujourd'hui l'objectif de 7 000 places livrées à l'horizon 2022.

Sur ce programme, la commission des lois a émis un avis défavorable. J'évoquerai maintenant l'aide juridictionnelle, un sujet qui me tient à coeur et sur lequel Jacques Mézard et moi-même avons été corapporteurs d'une Les moyens mobilisés devraient augmenter de 7 %, pour atteindre 507 millions d'euros. C'est une excellente chose, mais, au regard des contraintes pesant sur le budget de l'État, il sera vraisemblablement nécessaire de conforter ces financements.

Au-delà de ces aspects budgétaires, il est impossible de ne pas dire quelques mots sur la réforme de la justice, que j'évoquais à l'instant. Pour la discussion de cette réforme, essentielle pour notre République et les droits de nos concitoyens,

Il est pratique de bénéficier d'une majorité large et facile de se passer du concours de la deuxième chambre ; c'est aussi éminemment dangereux. Contre-pouvoirs et corps intermédiaires sont à la base de nos principes démocratiques. Ce texte est une catastrophe. On ne peut ignorer l'indignation unanime des professionnels du droit. Avocats et magistrats se sont mobilisés jeudi dernier pour une journée « justice morte ». Sinistre présage ... Syndicats, bâtonniers et avocats continuent d'être très actifs auprès de nous et, à titre personnel, je partage sans réserve leur profonde inquiétude.

Pour autant, cette augmentation est-elle suffisante pour adapter notre justice aux évolutions sociétales ? Vraisemblablement non.

Oserai-je ajouter que l'administration et l'exécutif sont peuplés de publicistes, mais que la justice nécessite aussi une vision de civiliste et de pénaliste et qu'il est utile d'écouter et de lire les observations et propositions émanant de la Cour de cassation.

et il n'est pas sain de considérer que l'on peut pallier cette carence simplement par la déjudiciarisation. Notre justice souffre de plusieurs maux. L'un des plus graves est la non-exécution ou l'exécution partielle des peines. Comment comprendre que des peines ne soient jamais exécutées, ou qu'elles le soient parfois des années après leur prononcé ? Voilà une vraie priorité pour une politique judiciaire. L'état de nombre de nos prisons en est une autre, surtout quand la prison fabrique de la récidive et des terroristes. Elle ne peut répondre à sa mission première, et la mise en place de peines alternatives

Je ne suis pas opposé- je ne l'ai jamais été -à une organisation départementale des juridictions, mais j'attire votre attention sur l'impérieuse nécessité de maintenir des juridictions à compétence généraliste. Continuer à spécialiser des juridictions dans quelques métropoles est une fausse bonne idée qui éloigne le justiciable de la justice et contribue à vider les territoires de la matière grise professionnelle.

la haute administration continuera à vouloir imposer une restructuration centrée sur ces grandes métropoles parce que cela l'arrange, l'État accentuera la fracture territoriale et sociale, dont nous constatons les dégâts cruels aujourd'hui. Il en est de même en ce qui concerne le système pénitentiaire. Je pourrais citer un certain nombre d'exemples aberrants de prisons à moitié vides parce que cela dérange l'administration d'y envoyer des détenus

Je persiste à dire qu'il y a d'autres solutions que recourir au budget de l'État. En particulier, les bénéfices réalisés par les compagnies d'assurances sur la protection juridique doivent être davantage sollicités pour financer l'aide juridictionnelle. C'est un choix politique fort à assumer

Christiane Taubira, qui voulait supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs créés sous Nicolas Sarkozy et donner la priorité aux mesures éducatives sur les mesures répressives.

Vous le savez, conformément au principe de la légalité des délits et des peines, les parents d'enfants délinquants peuvent être poursuivis sur le fondement de leur défaillance propre, qui constitue alors le fait générateur d'une infraction autonome. L'article 227-17 du code pénal punit en effet de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende « le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur Le texte existe, il est même plutôt bien rédigé, mais, dans les faits, les juges sont démunis. Les stages dits « de responsabilité parentale parentale », par exemple, faute d'associations en mesure de les mettre en oeuvre, ne peuvent être mis en place sur l'ensemble de notre territoire, ce qui crée des inégalités inadmissibles entre justiciables d'un département à l'autre. La mise en oeuvre des décisions de nature civile appartient certes aux départements. Cependant, nous le savons, ces derniers sont débordés par leurs missions, notamment par la prise en charge des mineurs étrangers isolés, dont le nombre a triplé depuis 2015.

je vous encourage à en réduire le nombre, afin que notre arsenal ne soit composé que de mesures applicables et appliquées. L'enjeu est très important

sociaux. Enfin, les différentes restrictions budgétaires rendent les recrutements difficiles. Les greffiers, en nombre insuffisant, peinent à remplir leurs missions.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues,

Monsieur le président, madame le ministre, universitaire, j'ai enseigné le droit toute ma vie professionnelle. Vous pouvez deviner combien les valeurs de la justice ont imprégné mes réflexions. Directeur de l'Institut d'études judiciaires de Lille, j'ai formé tous les ans des centaines d'étudiants, devenus par la suite avocats ou magistrats. Je leur disais très souvent : « N'oubliez pas que vous allez recevoir dans vos cabinets des personnes qui souffrent et et qui attendent de la justice une écoute, une prise en charge, de la compassion pour leurs problèmes familiaux ou professionnels, une réponse pénale à l'atteinte qu'ils ont subie sur leurs biens ou sur leur personne

Les tribunaux de grande instance, déjà en sous-effectif, vont devoir absorber dès janvier le contentieux social, qui était jusqu'à présent traité par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité,

Je ne peux que noter que nos concitoyens les plus fragiles n'ont pas obtenu la protection qu'ils étaient en droit d'attendre dans la programmation pour 2019. Je nourris de grandes craintes quant à l'évolution de la protection des personnes sous tutelle, des femmes victimes de violences et, surtout, des enfants en danger. par exemple, quelque 200 mineurs en danger ne peuvent être admis dans les structures d'accueil, faute de place. Des assistantes sociales, des médiateurs, des psychologues prennent en charge l'assistance éducative, que la loi confie pourtant confie pourtant au juge des enfants, aujourd'hui surchargé de travail. Pour moi le juge reste le juge, celui qui exerce l'autorité, qui a la responsabilité d'incarner la justice. La déjudiciarisation ne me semble pas répondre aux attentes des justiciables et au besoin d'une justice forte.

et la création de 1 300 emplois. Je remercie d'ailleurs le rapporteur spécial Antoine Lefèvre d'avoir souligné que cette augmentation était significative et équilibrée.

de budget que je vous présente traduit plusieurs priorités qui visent à assurer une transformation en profondeur de la justice. La première priorité est l'amélioration de la justice au quotidien.

tribunal d'instance ne fermera nulle part dans notre pays, car ma seule ambition est de maintenir cette justice de proximité au plus près de nos concitoyens.

même que, lorsque des besoins apparaîtront, de nouveaux contentieux puissent y être jugés. Tout cela sera garanti, je ne peux donc pas comprendre que l'on dise que les tribunaux de proximité fermeront : c'est inexact

de livrer 7 000 places de prison et d'engager la construction de 8 000 autres d'ici à 2022. Faisant cela, je ne ne présente pas un budget trompeur, pour reprendre l'expression que vous avez employée, mais un budget volontariste, soutenant une politique réaliste.

équilibrée, de nature à répondre à la pluralité des demandes des magistrats. En 2019, cette orientation se traduira notamment par le lancement du programme de construction de vingt centres éducatifs fermés, dont le nombre total sera ainsi porté à soixante ainsi porté à soixante et onze. Cela ira de pair avec l'augmentation du recrutement de familles d'accueil et le développement d'une plus grande pluridisciplinarité de l'intervention en milieu ouvert.

comme des professionnels, à procéder à la révision de l'ordonnance de 1945. C'est un texte qui a été modifié à de nombreuses reprises et qui, aujourd'hui, n'a plus de cohérence.

La dernière de mes priorités est de porter une attention particulière à nos concitoyens les plus vulnérables, grâce à une politique renforcée d'accès au droit et d'aide aux victimes. Les moyens consacrés à l'accès au droit et à la justice progressent de 6,5 % dans le budget pour 2019 pour atteindre 467 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 83 millions d'euros de ressources affectées, destinées au financement de l'aide juridictionnelle. Ce sont plus

l'action conduite par la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, placée à mes côtés, me semblent garantir que les victimes puissent bénéficier, sur la durée, d'un suivi dans les domaines psychologique, social et économique. Il faut conclure,

Monsieur le président, mon intervention se fonde non seulement sur le règlement, mais aussi sur la Constitution. Il se trouve qu'il y a deux assemblées dans le Parlement.

affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité au ministère de la justice. Cette réforme est mise en oeuvre grâce à un transfert des personnels relevant des organismes de sécurité sociale et du ministère

Compte tenu de la possibilité laissée aux agents relevant du ministère de la santé ou des caisses primaires d'assurance maladie de ne pas rejoindre le ministère de la justice, il est apparu que le nombre de 541 agents mis à disposition du ministère ne serait pas atteint. En conséquence, le projet de loi de finances transfère des emplois à hauteur de 84 équivalents temps plein pour permettre au ministère de la justice de recruter les personnels nécessaires au fonctionnement de ces pôles sociaux. Sur ces 84 emplois, 54 sont transférés depuis le ministère des solidarités et de la santé par un transfert de crédits et d'emplois du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » vers le programme « Justice judiciaire » et 32 emplois sont transférés depuis la sécurité sociale par une mesure de périmètre. Toutefois, au regard des nouvelles évolutions des effectifs qui seront effectivement présents au 1 janvier 2019 au sein des pôles sociaux, le nombre de 84

de la masse salariale du programme 166, à hauteur de 1 235 912 euros. Ce transfert complémentaire est indispensable à la bonne mise en oeuvre des réformes des juridictions sociales au 1 janvier prochain.

destinés au financement de l'aide juridictionnelle. Cette aide concerne près de 1 million de personnes, et le filtre permettant d'apprécier la recevabilité de la requête prévu par la loi de juillet 1991 n'est jamais mis en oeuvre.

et Jacques Mézard intitulé « Aide juridictionnelle, le temps de la décision ». Elle l'a fait de nouveau en 2017, au travers du rapport de la mission d'information sur le redressement de la justice. Sur sa proposition, le Sénat a introduit dans le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice des mesures concrètes et utiles pour réformer en profondeur l'aide juridictionnelle. J'y ai fait référence dans la discussion générale. L'inertie du Gouvernement est particulièrement regrettable, dès lors que le diagnostic et les pistes de réforme sont connus. C'est pourquoi, tout en partageant les préoccupations de mes collègues, je m'interroge sur l'utilité d'abonder sans fin les crédits de l'aide juridictionnelle, au détriment d'autres actions de l'autorité judiciaire, si ces majorations ne s'accompagnent d'aucune réforme structurelle. L'aide juridictionnelle ne doit pas devenir le tonneau des Danaïdes de la justice Quel est l'avis du Gouvernement ? Monsieur Mézard, vous proposez d'accroître les ressources extrabudgétaires qui financent l'aide juridictionnelle,

porté à 1 000 euros. Ces crédits permettront également de financer les conséquences de l'extension de la représentation obligatoire, prévue dans la loi de programmation et de réforme pour la justice. À ce stade, nous n'avons donc pas besoin de ressources financières supplémentaires.

pour un effet budgétaire en 2020. J'ai confié une mission aux inspections générales de la justice et des finances pour travailler sur des pistes concrètes d'amélioration du dispositif d'aide juridictionnelle. Ce rapport m'a été remis, et nous allons maintenant pouvoir travailler sur les pistes proposées,

je veille à ce que des réponses leur soient apportées, et je vous présente mes excuses si tel n'a pas été le cas pour le courrier que vous m'avez adressé.

Évidemment, les subventions versées par l'administration pénitentiaire vont à des associations qui participent au service public pénitentiaire, conformément à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 novembre 2009 ; nous devons collectivement justifier de leur bonne utilisation. Le ministère est lié de très longue date au GENEPI. Ce groupement, créé par Lionel Stoléru en 1976, a pour finalité de développer les contacts entre les étudiants de l'enseignement supérieur, souvent issus de grandes écoles, et le monde pénitentiaire. L'activité principale de l'association était jusqu'ici de donner, bénévolement, des cours aux détenus incarcérés.

en échange d'un engagement de l'association de stabiliser le nombre d'heures d'activité assurées au bénéfice des personnes détenues. Plusieurs éléments m'ont conduite à envisager le non-renouvellement de cette convention et de cette subvention.

Ce désengagement correspond en réalité à une évolution des missions que le GENEPI se donne au niveau national. En effet, l'association a retiré de ses statuts la mention

le GENEPI a adopté un positionnement très critique à l'égard de l'administration pénitentiaire, comme en témoigne le mot d'ordre d'un certain nombre de ses actions : « L'État enferme, la prison assassine ».

prévoit le développement, contribuaient à une « aliénation » des personnes détenues. Dans ces conditions, il nous est apparu qu'un financement public par l'administration pénitentiaire de l'activité du GENEPI était difficilement envisageable. Néanmoins, au regard de l'ancienneté de notre partenariat avec cette association, j'ai souhaité qu'un nouveau conventionnement, sans financement, puisse lui être proposé, afin de permettre aux étudiants qui le souhaiteraient de poursuivre leur activité d'éducation populaire en détention et d'avoir accès aux établissements pénitentiaires. Des dialogues sont en cours en ce sens entre mes services et le GENEPI.

Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Justice », figurant à l'état B. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix ces crédits, modifiés.

à l'exclusion des actes de notaire, des actes d'huissier de justice et des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ouvrent un droit proportionnel ou progressif. Ce dispositif est avantageux à double titre, du fait de son assiette large et de son taux bas. Il permet en outre de maintenir un lien entre la taxation proposée et ses futurs bénéficiaires. En se référant au tableau récapitulatif « Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes » du tome I du fascicule « Évaluations des voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2018, le produit résultant de l'augmentation de 1 % de ces droits s'élèverait à 180 millions d'euros, soit une somme nettement supérieure aux recettes extrabudgétaires de nature fiscale figurant, à hauteur de 83 millions d'euros, dans le présent

une période récente. Cette mesure a d'ailleurs été adoptée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cette démarche nous paraît plus pertinente que la création ou l'augmentation de diverses taxes affectées. J'ajoute que, pour des raisons de recevabilité financière, ces amendements tendent à augmenter des taxes

a abaissé le plafond de l'aide juridictionnelle à 1 000 euros pour une aide juridictionnelle totale et à 1 525 euros

perçus sur les actes juridiques mentionnés à l'article 635 du code général des impôts ne financent pas, aujourd'hui, l'aide juridictionnelle. Les droits d'enregistrement sont à titre principal affectés

... Il y a là une possibilité tout à fait certaine de financer en partie l'aide juridictionnelle, même si cela ne plaît pas du tout à Bercy,